mes chers collègues, je n'ai que du bonheur à être avec vous ce matin pour la dernière séance de l'année 2022. Je suis sûr que vous prendrez ensuite quelques jours de congé bien mérités.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

Nous considérons pour notre part que cette séquence budgétaire aura affaibli le pouvoir parlementaire. Certes, l'usage du 49.3 est constitutionnel, mais l'abus du 49.3 mine le parlementarisme et, dans le même temps, la confiance de nos concitoyens. Le Président de la République déclarait au soir du deuxième tour de l'élection présidentielle : « Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. N'oublions pas ces paroles et mesurons bien les dangers politiques nourris par le mépris du Parlement, ainsi que les doutes profonds qu'expriment régulièrement nos compatriotes. Acte

portant sur la proposition de loi visant à rétablir l'équité territoriale face aux déserts médicaux et à garantir l'accès à la santé pour tous, Mme Guylène Pantel souhaitait voter pour.

du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de finances pour 2023, considéré comme adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution (projet

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les sénateurs, l'année qui s'achève a été celle d'un choix d'une constance absolue : refuser que le choc d'inflation ne mette au tapis l'économie française. Depuis le premier jour, nous avons affirmé une ligne extrêmement claire, celle du soutien et de la protection. Protéger encore et protéger toujours : protéger les ménages, protéger les entreprises, protéger nos collectivités. Le projet de loi de finances que nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture, tout comme la loi de finances rectificative promulguée le 1 décembre dernier, resteront comme les textes des engagements tenus vis-à-vis des Français. Grâce aux mesures que nous avons proposées, la France est le pays d'Europe dans lequel les ménages sont les moins exposés à la flambée des prix. Ce rempart contre la vie chère, nous avons pu l'ériger parce que nous avons collectivement fait le choix d'un soutien public franc et massif. Une analyse de la direction générale du Trésor, publiée la semaine dernière, montre que l'État a pris à sa charge plus de la moitié du choc inflationniste et du choc énergétique que subit notre pays depuis plus d'une année. Entre le bouclier tarifaire que nous avons été les premiers à mettre en oeuvre en Europe, la ristourne sur les prix à la pompe, le chèque exceptionnel et la revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales, ce sont près de 110 milliards d'euros d'argent public qui ont été mis sur la table pour protéger les Français et notre économie. Ces mesures ont conduit l'État à assumer 52 % de la perte de revenus réels liée au choc énergétique, laissant les entreprises en assumer 42 % et les ménages 6 %. 6 %. Ce reste à charge de 6 % pour les Français, en des temps d'inflation, c'est évidemment trop : je n'ignore rien des difficultés de ces millions de ménages qui vivent à l'euro près. Toutefois, je vous le dis, mesdames, messieurs les sénateurs, nous pouvons être fiers d'avoir, en France, fait le choix de la protection. Nous avons choisi de protéger le pouvoir d'achat. Nous avons choisi de soutenir les Français et nos entreprises. Nous avons choisi de préserver au maximum l'activité économique et la croissance. Oui, une fois encore, nous avons fait le choix de la protection : c'est non seulement mais aussi un choix d'efficacité. Cette stratégie est efficace, car il vaut mieux investir pour préserver que payer pour réparer. Comme durant la crise sanitaire, notre pays a ainsi évité l'explosion de la pauvreté qui frappe certains de nos voisins européens. Cela a été possible notamment grâce à la revalorisation anticipée des prestations sociales dès l'été 2022, au financement d'une aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros pour 11 millions de familles, au versement d'un chèque énergie exceptionnel à 12 millions de ménages à la mise en place de dispositifs spécifiques pour nos concitoyens qui se chauffent au fioul ou au bois. En parallèle, notre politique en faveur du travail et de la stabilité fiscale continue de porter ses fruits, puisque le chômage se maintient à un niveau historiquement bas- 7,3 % -, tandis que l'investissement des entreprises résiste,

grâce aux millions d'entrepreneurs qui continuent d'investir et d'embaucher et grâce aux Français qui continuent autant que possible de consommer, parce que nous prenons des mesures pour protéger leur pouvoir d'achat. Le budget que nous présentons pour l'année prochaine traduit la continuité de cette stratégie, sans jamais perdre de vue que l'argent public, c'est l'argent des Français et que chaque euro investi doit être un euro efficace. Nous l'assumons : ce projet de loi de finances est un texte de combat contre la vie chère, qui prévoit le maintien des boucliers tarifaires et l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu.

le sentiment que l'argent public sert davantage à accompagner certains de nos concitoyens qui ne travaillent pas plutôt qu'à les soutenir eux, eux qui se lèvent le matin pour aller travailler. Il est extrêmement important que nous nous adressions aussi à ces Français qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui font des efforts dans un contexte et dans des circonstances parfois difficiles. Nous devons leur montrer que l'action et l'argent public sont aussi là pour eux.

C'est pour les Français qui travaillent que nous avons fait le choix de rehausser de 50 % le plafond du crédit d'impôt pour les frais de garde d'enfants, qui sera porté à 3 500 euros. C'est pour les Français qui travaillent et pour nos entrepreneurs que nous avons fait le choix de relever le plafond permettant de bénéficier du taux réduit d'impôt sur les sociétés pour les C'est pour les Français qui travaillent que nous avons fait le choix de redonner de l'oxygène à nos agriculteurs, avec la prorogation jusqu'à 2025 de la déduction pour épargne de précaution, ainsi que son indexation sur l'inflation. Ce projet de loi de finances, c'est aussi celui du réarmement de nos services publics. Ce texte donne plus de moyens à la police, à la justice et à nos armées dans un contexte géopolitique à haut risque.

Enfin, nous poursuivons le renforcement des moyens du ministère de la justice, avec une nouvelle hausse des crédits de 8 % pour la troisième année consécutive. Au total, depuis 2017, la hausse des crédits du ministère de la justice justice a été de 40 %. Si nous agissons pour lutter contre l'insécurité, nous agissons aussi pour lutter contre l'impunité et pour faire en sorte que notre justice puisse fonctionner plus efficacement et plus rapidement. Tout cela s'inscrit en cohérence avec le choix que nous avons fait dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale 2023. L'an prochain en effet, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le budget de l'hôpital public dépassera les 100 milliards d'euros. En matière économique, notre principal objectif est de gagner la bataille du plein emploi d'ici à 2027. C'est grâce au travail des Français que la croissance résiste. C'est par l'augmentation du volume de travail que nous serons en mesure de créer plus de richesses et de les redistribuer. Le plein emploi commence par l'éducation. L'année prochaine, le budget de l'éducation nationale augmentera de près de 4 milliards d'euros : comme le Président de la République s'y était engagé pendant la campagne, aucun professeur ne commencera sa carrière inférieur à 2 000 euros net par mois. Le plein emploi, c'est aussi l'apprentissage. Quelque 6,7 milliards d'euros de crédits supplémentaires seront investis dans l'emploi et l'apprentissage pour atteindre l'objectif du million d'apprentis d'ici à 2027. Enfin, et je le dis avec fermeté, ce texte acte le refus catégorique du laisser-aller budgétaire. Comme ministre chargé des comptes publics, je continuerai de défendre le « combien ça coûte », parce que l'argent public ne sera jamais de l'argent magique. Oui, malgré les aléas, nous poursuivons le rétablissement des comptes amorcé dès 2021, en stabilisant le solde public à 5 % cette année, comme en 2023. Nous y parviendrons parce que nous maîtrisons l'évolution des dépenses. Nous y parviendrons aussi grâce aux recettes liées à la contribution sur les rentes inframarginales. dernier, nous évoquions notre volonté de nous inscrire dans un cadre européen, certains ont cru y voir une manoeuvre dilatoire, une façon de balayer le problème d'un revers de la main. La réalité, c'est que nous ferons entrer 11 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État, l'année prochaine, grâce à cette contribution sur les rentes inframarginales des énergéticiens. Ils permettront de financer nos mesures en faveur des ménages, des entreprises et des collectivités locales. Ces grands objectifs, nous avons eu l'occasion d'en discuter de manière approfondie. le débat a également permis d'enrichir significativement le texte qui vous est aujourd'hui présenté. Bon nombre d'ajouts issus de cette assemblée ont été retenus dans la version finale du texte. Je ne peux pas être exhaustif, mais vous me permettrez de mentionner un certain nombre de mesures.

Je pense à l'introduction de crédits d'impôt, pour les entreprises comme pour les particuliers, sur les dons aux communes et syndicats forestiers pour certaines opérations de gestion forestière. Le sujet, mis en avant notamment par Vanina Paoli-Gagin et par le groupe Les Indépendants, était d'ailleurs au coeur d'une proposition de loi adoptée en première lecture dans cet hémicycle. Je pense à l'établissement d'une base légale à l'exonération d'impôt dont bénéficient déjà les allocations versées aux orphelins de victimes d'actes antisémites et d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, sur l'initiative de Marc Laménie, qui a déposé cet amendement. Sur nos outre-mer, nous avons également intégré plusieurs amendements importants. Je pense à l'amendement du rapporteur général de la commission des finances visant à inclure les collectivités d'outre-mer dans le périmètre des dispositifs de défiscalisation prorogés. Je mentionne également la prolongation de plusieurs dispositifs de défiscalisation jusqu'en 2029

Concernant la Corse, nous avons retenu dans le texte deux amendements défendus par Jean-Jacques Panunzi : l'un prévoit la prorogation du crédit d'impôt en Corse jusqu'en 2027, l'autre permet de garantir l'éligibilité de ce même crédit d'impôt aux résidences de tourisme.

Bon nombre de mesures sont d'ailleurs, directement ou indirectement, le résultat des échanges que nous avons eus et des compromis que nous avons su construire malgré un certain nombre de désaccords légitimes, je le crois, en démocratie.

ajoutée des entreprises (CVAE), nous garantissons une compensation à l'euro près avec une fraction pérenne de TVA. La compensation sera calculée en faisant une moyenne sur quatre années, de 2020 à 2023. Je sais que cela constituait une préoccupation forte à ce que les bonnes années en matière d'activité économique, en d'autres termes les toutes dernières années, puissent être prises en compte dans ce calcul. Quant au filet de sécurité, il sera étendu à l'ensemble des strates de collectivités, en l'espèce, les départements et les régions. Cette version de 2023, largement inspirée par les travaux du Sénat, a été remaniée de la façon suivante : nous supprimons le premier critère d'éligibilité ; le seuil de perte d'épargne brute est fixé à

Comme vous le savez, notre soutien se poursuivra l'année prochaine pour aider les communes à faire face à la flambée des coûts de l'énergie. Le dispositif des tarifs réglementés d'électricité en 2023 pour les petites communes est complété par un amortisseur électricité qui s'appliquera dès le 1 janvier. Concrètement, cela signifie que les collectivités territoriales qui ne sont pas éligibles au bouclier tarifaire seront également soutenues par l'État, et ce quelle que soit leur taille : pour un tarif entre 180 euros et 500 euros le mégawattheure, nous prendrons en charge la moitié de leur facture d'électricité.

J'espère que, au Sénat, ce débat se déroulera toujours dans le même esprit de dialogue respectueux de nos institutions, respectueux de la courtoisie républicaine, respectueux- je le crois profondément -des attentes des Français, qui souhaitent que nous nous parlions et que nous travaillions ensemble. Monsieur le

En effet, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie le 6 décembre dernier, n'a pu aboutir favorablement, en raison de la persistance de divergences trop importantes portant sur les 237 articles restant en discussion. Notons qu'en première lecture l'Assemblée nationale et le Sénat avaient déjà adopté, dans les mêmes termes, 88 articles. À l'issue de la nouvelle lecture, le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale- qui est finalement le vôtre, monsieur le ministre -a parfois suivi le Sénat, même partiellement. J'en présenterai quelques exemples, avant de vous indiquer, toutefois, les nombreux désaccords qui demeurent entre nos deux chambres.

Celui-ci consistait, en réalité, à réintroduire le dispositif de contractualisation et de sanction, souhaité par le Gouvernement, à destination des collectivités territoriales, alors même que celui-ci avait été rejeté par les deux assemblées lors de l'examen du projet de loi de programmation des finances publiques

Plusieurs mesures de prorogation ou d'amélioration de dépenses fiscales assurent un soutien, notamment économique ou dans la lutte contre l'habitat indigne, aux collectivités d'outre-mer, qui font face à des contraintes et à des difficultés spécifiques. Il en est de même pour la Corse. Je me réjouis aussi du maintien, non pas de tous, mais de plusieurs dispositifs visant à lutter contre la fraude fiscale, qui constituent la traduction législative de recommandations issues l'évasion fiscales, créée par la commission des finances. Je salue également le fait que le texte reprenne la position du Sénat en conservant, sous réserve de divers aménagements, l'essentiel des modifications apportées à la nouvelle contribution sur la rente inframarginale, applicable aux producteurs d'électricité. Pour autant, sur les mesures fiscales et budgétaires relatives à l'énergie, je rappelle que le Sénat a fait preuve d'un sens aigu

conformément aux décisions prises à l'échelon européen. En effet, je le rappelle, monsieur le ministre, nous avons accepté de voter des dispositifs qui n'ont cessé d'évoluer de façon majeure au cours de la navette parlementaire, sans que nous ayons pu disposer d'études d'impact suffisamment solides ni même de tous les éléments nous permettant de comprendre parfaitement l'ensemble des enjeux des modifications opérées.

Pour autant, malgré le maintien de ces apports du Sénat, des désaccords importants subsistent entre les positions de notre assemblée et celles qui figurent dans le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale, sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité.

Quand la dette publique atteint 111,5 % du PIB, la remontée des taux d'intérêt constitue un risque pour la soutenabilité de notre dette. S'il est vrai que l'inflation est mieux maîtrisée en France que dans d'autres économies développées, c'est au prix d'une forte mobilisation

le budget de l'État, le Gouvernement fait en réalité le choix d'identifier les dépenses qui doivent continuer à augmenter, sans s'occuper des économies qui devraient les compenser. Ce n'est pas faire preuve de responsabilité. Le déficit de l'État, supérieur à 150 milliards d'euros pour la quatrième année consécutive, reste sur les sommets atteints pendant la crise sanitaire. Ce budget est celui de tous les records en termes de niveau, aussi bien de déficit présenté en loi de finances initiale que d'emprunts nouveaux.

(CVAE), est opéré sans que soient proposées de meilleures garanties quant aux modalités de compensation prévues pour les collectivités territoriales. Pourtant,

tenant compte de l'inflation ou encore de la prorogation, pour une année supplémentaire, du renforcement du crédit d'impôt pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire. Je reviens aux finances locales. réjouir du fait que, sous la pression du Sénat et du dispositif que nous avions adopté, le Gouvernement ait été contraint d'ouvrir davantage les conditions d'éligibilité au filet de sécurité prévu pour les collectivités territoriales et je le regrette -, la conservation du critère de perte d'épargne brute, même réduit à 15 %, est une mauvaise nouvelle pour deux raisons : d'une part, il est fortement excluant et générateur d'importants effets de seuil ; d'autre part, il ne me paraît pas utile pour s'assurer que les collectivités doivent être aidées, dans la mesure où les modalités mêmes de calcul de la dotation mettent déjà en relation la différence entre la progression des dépenses et celle des recettes. Notre proposition, qui visait à rendre éligibles un plus grand nombre de collectivités territoriales durement touchées par la crise, donc à étendre la protection qui leur serait apportée, était à mon sens à la fois juste, équitable et raisonnable.

Je ne comprends pas non plus pourquoi la majorité gouvernementale ne nous a pas rejoints autour d'amendements pourtant votés à la quasi-unanimité. Ainsi en est-il du relèvement du plafond du prêt à taux zéro qui doit permettre de soutenir l'accession à la propriété des primo-accédants, sous conditions de ressources, dans un contexte de durcissement des conditions d'emprunt immobilier. Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale a également rétabli les crédits des quatre missions qui avaient été rejetés par le Sénat, sans apporter aucune réponse aux objections du Sénat.

déjà la confirmation que le Gouvernement s'est bien ménagé une confortable réserve de crédits au sein de la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles (DDAI). En effet,

Ces crédits, tels qu'ils étaient inscrits dans le texte initial, avaient donc une tout autre destination. Cela n'est évidemment pas satisfaisant pour le législateur. Monsieur le ministre, vous le constatez, les sujets de désaccords entre le Sénat et la

Que reste-t-il de nos 160 heures de débat et, encore plus, du travail effectué en amont et en commission ? Sans surprise, le Gouvernement est revenu sur l'amendement de la majorité sénatoriale prévoyant un dégrèvement de la CVAE pour les entreprises plutôt que sa suppression sèche. La suppression en deux ans de cet impôt territorial est une mesure emblématique du budget 2023. Nous resterons attentifs aux modalités de compensation, annoncées à l'euro près, à destination des collectivités territoriales. Les contributions exceptionnelles sur les bénéfices des entreprises du secteur de l'énergie entreront également en vigueur, bien que des modifications techniques et relatives à leur périmètre puissent encore être apportées- le diable est dans les détails.

sur les services numériques, mise en place en 2019, qui avait attiré le courroux de nos partenaires d'outre-Atlantique. Quoi qu'il en soit, l'exécution du budget 2023 sera cruciale. Elle dépendra plus que jamais de l'évolution de la conjoncture macroéconomique. Espérons qu'elle sera plus favorable que ne l'affirment certains prévisionnistes, parfois un peu alarmistes, alors que le coût des intérêts de la dette publique a explosé en 2022.

la taxe d'aménagement, la suppression de la réforme de la répartition au sein du bloc communal, votée l'an dernier, nous paraît préférable, dans la mesure où les charges d'aménagement varient fortement en fonction de chaque territoire.

En conclusion, les membres du groupe RDSE, attachés à la poursuite du débat parlementaire, s'opposeront, sur la forme, à la motion tendant à opposer la question préalable, même s'ils en comprennent les motivations.

Monsieur le ministre, la déception est forte. Tout ça pour ça ! Après 160 heures de séance au Sénat, l'examen de plus de 3 000 amendements et l'adoption de plus de 600 d'entre eux, très peu d'apports de la Haute Assemblée ont été finalement Le Gouvernement, une nouvelle fois, fait peu de cas du Parlement. Nous sommes pourtant la seule chambre qui, cette année, a examiné l'ensemble du texte. Nous vous avons fait des propositions constructives. Quasiment tout a été balayé, y compris les mesures adoptées à la quasi-unanimité du Sénat, comme le prêt à taux zéro ou la limitation des bonus pour les véhicules électriques. Mes chers collègues, je salue notre travail collectif tout au long de la discussion, malgré quelques moments curieux, et l'action de notre rapporteur général, toujours efficace et bienveillante, avec pour seul souci l'intérêt général. Pourtant, vous prétendez qu'une méthode nouvelle devait être mise en place et vous ne cessez de demander à chacun, à la droite républicaine en particulier, de travailler avec vous, dans l'intérêt du pays. En réalité, la main que vous tendez est un poing fermé. À quoi bon perdre son temps dans les pseudo-dialogues de Bercy, ou même dans nos débats, pour en arriver à ce déni total de notre régime parlementaire ? Vous ne voulez pas écouter, alors même que, comme nous l'avions dénoncé dans la discussion générale, votre budget est l'un des pires jamais présentés, loin d'une gestion à l'euro près.

Je veux toutefois ouvrir une parenthèse pour vous remercier, monsieur le ministre, de votre présence et de vos réponses, même si vous ne nous avez finalement pas entendus, ce qui risque de rendre le dialogue plus difficile demain. Que le Gouvernement se dessaisisse de la question de la réduction de la dépense, dans le contexte de l'envolée de notre dette, en disait déjà beaucoup sur son manque de responsabilité. Qu'il ne reprenne finalement aucune de nos propositions d'économies, alors même qu'il nous avait mis au défi de lui en proposer, montre que, encore une fois, tout cela n'était que de la communication. Les calculs politiques semblent plus importants que l'intérêt du pays. Nous avions pourtant proposé 4,3 milliards d'euros d'économies, conformément à la trajectoire que nous avions votée dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années Il en est de même des mesures que nous avions adoptées pour venir en aide aux entreprises et aux collectivités territoriales, confrontées à une explosion de leurs factures énergétiques,

prend de nouveau comme référence l'évolution des dépenses d'énergie entre 2022 et 2023, plutôt qu'entre 2021 et 2023, alors qu'il s'agit là du bon étalon de mesure.

en vertu duquel toutes les collectivités territoriales, sans critère aucun, percevaient une dotation égale à 50 % de la différence, si elle était positive, entre l'augmentation des dépenses d'énergie entre 2023 et 2021 et 40 % de la hausse de ses recettes réelles de fonctionnement sur la même période.

Pour ce qui concerne la territorialisation, les critères du nouveau fonds national d'attractivité économique des territoires ne sont toujours pas précisés : ils restent renvoyés à un décret ultérieur. Nous voterons donc ce dispositif à l'aveugle, ce qui est on ne peut

cette évolution de la CVAE, quoi qu'on en pense par ailleurs- vous savez que nous y sommes favorables sur le principe -, n'aura bénéficié d'aucune approbation parlementaire. Plus qu'un problème, c'est une alerte.

J'aurais pu citer bien d'autres exemples, mais le temps est compté. Si nos entreprises lâchent, victimes de la crise énergétique, c'est notre pays tout entier qui dévisse.

Nous le regrettons d'autant plus que ce texte contient des mesures importantes pour les collectivités territoriales. Nos élus locaux attendent un véritable soutien pour lutter contre l'inflation. Ces mesures sont à la fois fortes et nombreuses, à tel point que nous devons désormais faire un effort de pédagogie pour que nos collectivités puissent tirer profit des dispositifs qui seront mis en place en 2023. Entre les annonces égrenées par le Gouvernement pendant tout l'automne et les discussions parlementaires, les élus sont perdus. Ils ont besoin d'y voir plus clair sur ce qui figure finalement dans le texte. Nous prendrons notre part du travail nécessaire pour faire connaître ces dispositifs, mais la démarche doit être collective.

qu'il n'était à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale et plus restrictif que celui qu'a voté le Sénat : il s'agit donc d'une solution intermédiaire. Je remarque d'ailleurs qu'une perte d'épargne brute de 15 % correspond à ce que notre groupe avait proposé par la voie d'un sous-amendement à l'amendement de M. le rapporteur général. Ce critère permettra de couvrir la majorité des collectivités territoriales frappées par la hausse des coûts de l'énergie. Ce n'est pas une solution idéale, mais c'est une solution raisonnable. Elle ne résoudra pas toutes les difficultés des collectivités, mais elle limitera largement l'impact de l'inflation sur les finances locales. En outre, le filet de sécurité ne constitue que l'un des volets du mécanisme de soutien. Pour les plus petites communes, le bouclier tarifaire continuera de s'appliquer en 2023. Pour les communes qui ne seraient éligibles ni au bouclier tarifaire ni au filet de sécurité, il restera l'amortisseur électricité.

finances : si « leur épargne brute a enregistré, en 2023, une baisse de plus de 15 % [ ...] parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seul[es] sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée [ ...] les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales

Cet exemple illustre le traitement réservé à nos 160 heures de débat et aux quelque 3 000 amendements que nous avons discutés. Vous êtes dénué de majorité à l'Assemblée nationale, mais vous continuez à gouverner seuls, dans un entre-soi dangereux pour la démocratie et pour nos institutions. Vous avez fait votre « tri sélectif » parmi les amendements votés pour revenir, le 49.3, à la maquette à peine modifiée du texte initialement présenté à l'Assemblée nationale. Pour l'essentiel, vous avez retenu les amendements gouvernementaux

Certes, le 49.3 est constitutionnel. Évidemment, vous faites bien de ne pas laisser un texte qui supprime cinq missions budgétaires poursuivre son chemin. Pour autant, cela ne justifie pas de ne rien retenir, ou presque, de nos L'inutilité de nos débats et non-débats laisse trop de place au Rassemblement national, qui en profite pour apporter ses mauvaises réponses à de bonnes questions.

Vos déclarations publiques annoncent, hélas ! la poursuite des décisions jupitériennes, ignorant le Parlement comme vous ignorez les partenaires sociaux avec votre réforme néfaste des retraites. Monsieur le ministre, on a rarement raison seul. La démocratie sans Parlement et sans partenaires sociaux, ce n'est déjà plus la démocratie.

Avec l'amortisseur électricité et le filet de sécurité, la France dispose du système de protection le plus complet et le plus ambitieux déployé en Europe. Au cours de la navette parlementaire, le Gouvernement et les députés ont conservé des apports importants

En dépit de tous ces efforts pour protéger les Français et réarmer nos services publics, en dépit des nombreuses concessions faites, la majorité sénatoriale choisit de nous priver de ce débat ... Oh ! ... et de se dessaisir elle-même de sa responsabilité.

Il vous aura fallu improviser une seconde délibération portant sur un certain nombre d'amendements de la première partie pour afficher un déficit à peine en recul.

personnellement et individuellement, mais, tels les membres d'une équipe de foot qui perd, vous omettez de parler entre vous, d'agir collectivement et en cohérence sur le terrain, ... Très bonne image ! ... au point, très souvent, de procéder dans l'hémicycle à des votes en totale contradiction avec vos choix en commission.

Les élus, les partis politiques, la presse et les Français le font suffisamment pour que- je l'espère -vous mesuriez le poids de ces décisions sur la perception que notre nation a de ses politiques, de son gouvernement et de ses élus.

face à l'inflation galopante, la fraternité devrait être le maître-mot de l'action publique, vous tous avez fait le choix de vous obstiner en poursuivant sur la voie du libéralisme

de même pour les dépenses. En dépit de la mise en échec systématique de nos dispositions en matière de recettes, qui vous aurait donné des marges budgétaires supplémentaires, nous avons tenu à vous faire de nouvelles propositions. Malheureusement, force est de constater que le maintien des services publics dans les territoires, notamment ruraux,

mais votre budget sera adopté sans avoir été voté ... On ne gagne jamais contre la démocratie. Les administrations publiques, la sécurité sociale ou les collectivités territoriales sont confrontées à un gouvernement qui fuit ses responsabilités. Ce budget marque le désengagement de l'État sur le financement de la formation continue, le compte personnel de formation, au détriment des travailleurs, et sur le financement de l'apprentissage dans la fonction publique territoriale, au détriment des collectivités, En vérité, le partage de la valeur créée est sans cesse raboté et sans cesse volé aux travailleuses et aux travailleurs- en voilà un angle mort dans votre budget ! Partager la valeur, c'est pourtant accroître la contribution du capital, en mobilisant les transactions financières, les dividendes ou les bénéfices par exemple, mais c'est également s'interdire de faire payer les mesures de soutien aux ménages et aux collectivités par l'ensemble des concitoyens. Ensuite, vous créez une fiction : vous prétendez aider ceux qui subissent l'explosion des prix de l'énergie

la métropole du Grand Paris contre les établissements publics territoriaux, les communes rurales contre les communes urbaines, les départements selon leur potentiel financier, les autorités organisatrices de mobilités d'Île-de-France contre celles

mais attentif, en séance publique, où pas moins de 3 000 amendements ont fait l'objet de discussions, nous sommes réunis aujourd'hui pour nous prononcer sur le projet de loi de finances pour 2023 adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, après engagement par le Gouvernement de sa responsabilité sur le fondement de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. Nous vous le disons clairement, monsieur le ministre : nous regrettons qu'un aussi grand nombre de mesures adoptées par le Sénat n'aient pas été prises en compte par l'Assemblée nationale et le Gouvernement dans la version finale. Bruno Le Maire nous avait indiqué en ouverture des débats être « à l'euro près ». Visiblement, il n'est pas « au milliard près » ... Plusieurs mesures volontaristes de rationalisation des niches fiscales, en d'autres termes d'optimisation des ressources publiques, adoptées l'initiative du groupe Union Centriste, ont ainsi été balayées d'un revers de main par l'exécutif, sans la moindre explication, ni même parfois le moindre chiffrage de la part de Bercy. Les crises sont devenues omniprésentes. Il nous faut composer avec elles. Leur multiplication a pour inéluctable conséquence de détériorer la situation de nos finances publiques.

C'est dès 2023 qu'il aurait fallu engager les comptes de l'État sur la voie du redressement. Plusieurs amendements de notre groupe, qui une fois de plus aura eu le sens des responsabilités, y auraient contribué.

S'il est parfaitement légitime que la collectivité publique vienne au chevet des entreprises lorsqu'elles sont en difficulté, il est non moins légitime que ces mêmes entreprises, lorsque leur santé est meilleure, concourent à l'effort collectif d'assainissement des comptes publics. De même, la suppression de l'article 5, qui aurait sauvé la CVAE perçue par le bloc communal et les départements, aurait garanti à la sphère publique de sauvegarder immédiatement près de 4 milliards d'euros de recettes fiscales, tout en préservant l'autonomie financière des collectivités locales, malmenée depuis de trop nombreuses années. Eh oui ... Parmi les mesures adoptées pour soutenir nos collectivités territoriales figurait la réintégration dans le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) des opérations d'aménagement et d'agencement, qui y étaient devenues inéligibles du fait de la réforme de l'automatisation. Nous avions volontairement laissé de côté les opérations d'acquisition, par souci, là encore, d'en limiter le coût pour les finances publiques. Le Gouvernement n'a, hélas ! pas conservé la disposition du Sénat, pourtant légitime et nécessaire au regard des investissements élevés que les collectivités ont engagés. Par ailleurs, nous avions substantiellement simplifié et renforcé le filet de sécurité, pour le rendre accessible à un plus grand nombre de collectivités touchées par la crise énergétique, afin de leur permettre d'aborder plus sereinement les échéances à venir. Le Gouvernement lui-même semblait admettre la trop grande complexité des critères retenus dans le dispositif au titre de l'année 2022. Pour autant, que fait-il pour l'année 2023 après avoir recouru au 49.3 ?

Sans surprise, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 6 décembre dernier n'a pas été conclusive. Ainsi que l'a rappelé le rapporteur général, un trop grand nombre d'articles restaient en discussion. Compte tenu non seulement de l'échec de la commission mixte paritaire, mais également des délais prévus par la Constitution qui rendent impossible l'examen complet du texte en nouvelle lecture, le groupe Union Centriste adoptera quasi unanimement la motion tendant à opposer la question préalable. La discussion

à résoudre une équation évidemment complexe : tenir nos comptes et maintenir notre objectif de déficit à 5 %, tout en accompagnant les Français, les entreprises et les collectivités locales pour faire face au choc de l'inflation et de la hausse des prix de l'énergie

L'impôt n'est ni une injure ni un gros mot, monsieur le ministre, quand il est bien utilisé et qu'il permet de répartir correctement la richesse produite par les Français.

Le scrutin est ouvert.

portant sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, Mme Nathalie Goulet souhaitait voter contre. Acte